Pour ce faire, il faut simplement l'accord du maire de la commune d'accueil, sans que le maire de la commune de résidence ait son mot à dire. L'exercice de cette possibilité peut avoir des conséquences néfastes dans les communes rurales, puisqu'il conduit à diminuer les effectifs de l'école et peut aller jusqu'à menacer la pérennité de certaines classes et, parfois, de l'école elle-même.

il apparaît opportun que son inscription dans une école d'une autre commune soit subordonnée à l'accord du maire de la commune de résidence. Cette disposition ne concernerait que les communes de moins de 5 000 habitants et ne serait pas applicable dans les cas où l'inscription dans un établissement particulier est est justifiée par des motifs légitimes : contraintes professionnelles des parents, raisons médicales ou encore inscription dans le même établissement qu'un frère ou une soeur. Quel

particulières énumérées, la commune d'accueil ne recevra aucune participation financière de la part de la commune de résidence. Soumettre cette inscription à l'accord du maire de la commune de résidence lorsque celle-ci dispose d'une capacité d'accueil suffisante dans son école ne me semble pas la solution. Cela conduirait à une restriction

à la commune où est scolarisé l'enfant. Dans ce cas, les parents sont libres de choisir le lieu de scolarisation de leurs enfants. Or cette liberté de choix peut avoir d'importantes conséquences financières pour la commune de résidence, les frais de scolarisation variant sensiblement d'une commune à une autre. Ainsi, dans le département de l'Eure,

Ces frais peuvent ainsi représenter la totalité des recettes fiscales d'une commune et de l'ordre de 80 % de ses recettes totales. Aussi, il apparaît de bon sens que le maire puisse refuser l'inscription dans une école quand les frais de scolarisation sont moins élevés dans une autre école, située à une distance raisonnable de la commune de résidence. Ce droit de refus ne pourrait pas s'exercer dans les cas où l'inscription dans un établissement particulier est justifiée par des motifs légitimes : contraintes professionnelles des parents, raisons médicales ou inscription dans le même établissement qu'un frère ou une soeur. Quel monsieur le rapporteur.

Cette mesure de justice sociale doit en priorité profiter à ces enfants. Or l'accueil de tous les élèves âgés de 3 ans y sera matériellement impossible à la rentrée scolaire de 2019. Dans ce contexte, il semble indispensable de prévoir dans la loi un rapport rendant compte, au plus tard le 31 octobre 2021, de la mise en oeuvre de cette mesure.

Comme évoqué précédemment, la commission a supprimé l'article 7 , qui prévoyait un rapport sur le fléchage des financements perçus par Mayotte dans le cadre du plan Mayotte au titre de l'éducation des enfants non scolarisés, la structuration et la promotion dans le système éducatif des langues régionales à Mayotte et, enfin, l'application en Guyane et à Mayotte de l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire. Dans le prolongement de l'amendement n° 370 que nous venons d'examiner, cet amendement vise à récrire l'article 7 afin de circonscrire son périmètre

En effet, il existe dans l'enseignement des approches pédagogiques spécifiques aux milieux plurilingues dans certains territoires ultramarins, en particulier en Guyane. En revanche, Mayotte connaît un retard patent en la matière, le shimaoré

dans des conditions dérogatoires prévues par décret », en vertu de l'article L. 314-1. Des dérogations peuvent être apportées aux obligations légales pour procéder à des expériences pédagogiques, pour une durée limitée, avec la possibilité, pour les familles qui ne souhaitent pas y soumettre leurs enfants, d'avoir accès à un autre établissement, aux termes de l'article L. 314-2. Sous réserve de l'autorisation des autorités académiques et pour une durée limitée à cinq ans, les expérimentations peuvent porter sur des domaines cités par la loi : l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'utilisation des outils et ressources numériques, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. À mon sens, le projet de loi complète trop largement le champ de ces expérimentations, qui pourront désormais concerner la répartition des heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année, l'orientation, la liaison entre les différents niveaux d'enseignement, la participation des parents à la vie de l'établissement. À cette liste, notre rapporteur a souhaité ajouter l'enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale. Il est prévu d'associer les collectivités territoriales à la définition « des grandes orientations et des expérimentations menées par l'éducation nationale ainsi qu'à leurs déclinaisons territoriales certaines de ces expérimentations nous paraissent justifiées et intéressantes sur le plan pédagogique, d'autres, en revanche, nous semblent dangereuses. Il en va ainsi

Concernant les heures d'enseignement, on voit les limites de l'organisation hebdomadaire, qui empêche réellement l'innovation pédagogique des établissements. Pourquoi, par exemple, ne pas permettre un élève de quatrième d'avoir deux heures de musique toutes les deux semaines, au lieu d'une heure hebdomadaire perdue au milieu de son emploi du temps ? Pourquoi ne pas autoriser le renforcement du volume horaire en français et en mathématiques au début de l'année de sixième ? Plutôt que d'imposer des emplois du temps trop encadrés, il me semble qu'il faut donner aux établissements la liberté de les ajuster aux besoins de leurs élèves, à condition bien sûr qu'ils respectent le volume global prévu sur l'année. Cela permettra aussi de reconnaître que les professeurs ne sont pas que des exécutants, mais aussi des concepteurs de leur métier. les procédures d'orientation, la disposition prévue permettra aux établissements qui le souhaitent d'entrer dans l'expérimentation qui donnera le dernier mot à l'élève, prévue par la loi du 8 juillet 2013. L'ajustement du service des enseignants est donc une autre liberté

Pourtant, faute d'être présentée dès l'école comme une voie naturelle, la mobilité est parfois vue comme un pis-aller. De fait, certaines craintes concernant la coupure avec la famille s'épanouissent et empêchent, à l'âge adulte, les jeunes de franchir le pas. Il est donc vital que, dès le plus jeune âge, la mobilité soit vécue comme un enrichissement et une voie naturelle d'apprentissage ou de recherche d'un emploi. Cet amendement prévoit d'autoriser certains établissements pilotes à expérimenter des actions en ce sens.

je souhaite la suppression de cet alinéa.

introduite en commission, sur l'initiative de notre collègue Françoise Laborde, visant à donner aux familles la liberté de demander l'inscription de leur enfant dans un établissement ne pratiquant pas d'expérimentation. Cette garantie existe dans le droit en vigueur et n'a donné lieu, à ma connaissance, à aucune dérive. En conséquence, l'avis est défavorable.

toute famille qui le souhaite s'agissant d'une expérimentation approuvée par le conseil d'école ou le conseil d'administration, où les représentants des parents d'élève siègent me paraîtrait de nature à déstabiliser le fonctionnement de l'établissement. L'alinéa 8 permet aux familles qui le souhaitent d'inscrire leur enfant ailleurs, ce qui me semble une garantie suffisante. Avis défavorable.

il est précisé que l'article L. 111-1 du même code est applicable aux établissements d'enseignement privé qui sont associés au service public par contrat. Or ce dernier article définit les grands objectifs du service public de l'éducation, dont la mixité sociale. En outre, j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, ce sujet est au coeur des discussions que nous avons avec

ou externe de l'évaluation. Vous avez choisi de renforcer les capacités d'évaluation de votre ministère, c'est votre droit. Je trouve même légitime qu'un ministre se donne les moyens, en modifiant l'organisation de ses services, de renforcer certaines missions d'évaluation.

de ce projet de loi. Cet article reprend une préconisation de longue date du Sénat : l'évaluation des établissements scolaires. Le conseil d'évaluation de l'école reprendra l'essentiel

monsieur le ministre.

Monsieur Grosperrin,

et systémique, ce que mon collègue Grosperrin a traduit par « politique ». En effet, c'était une agence d'évaluation des politiques publiques en matière d'enseignement

qu'il pérennise cette chaire. Nous avons donc bien besoin de cet organisme extérieur d'évaluation systémique.

à Mme Sylvie Robert. Cet amendement tend à préciser les modalités de saisine du futur conseil de l'évaluation de l'école soit par autosaisine, soit par les ministres compétents, soit par les commissions compétentes des deux assemblées.

et des résultats de l'enseignement scolaire, il ne nous semble pas souhaitable de priver le nouveau conseil de l'évaluation scolaire de cette compétence de recherche et d'évaluation, alors même que nous avons besoin de repères précis quant à notre système.

qui vise à intégrer la mesure de la mixité sociale des établissements à tous les stades de l'évaluation, est en grande partie satisfait par le droit existant : un indice de position sociale des élèves, établi par la DEPP, permet de mesurer la composition sociale des classes et des établissements. Ces éléments seront pleinement pris en compte dans les évaluations d'établissement.

Et cela va mieux en le disant. L'amendement n° 340 rectifié a pour objet de s'assurer du caractère transversal et intégré de la transmission de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'enseignement scolaire, les missions du conseil d'évaluation de l'école. L'évaluation n'est pas qu'un outil formel de contrôle des connaissances. Elle s'exerce tout au long des enseignements et des contenus pédagogiques. Si elle vise bien évidemment à vérifier que les référentiels de compétences ont bien été acquis, elle s'assure également de la qualité de la transmission, afin d'adapter les contenus au quotidien et aux élèves. L'égalité entre les femmes et les hommes fait partie des valeurs qui doivent être transmises par l'école de la République. Cette volonté pédagogique étant relativement récente, il est difficile d'en quantifier les résultats concrets. Afin de renforcer l'effectivité de cette transmission, le présent amendement tend à intégrer aux missions du conseil d'évaluation de l'école le suivi de la transmission de l'égalité entre les femmes et les hommes. Madame Robert,

Mme Jacky Deromedi. Inspiré par les travaux du CEC, cet amendement vise à compléter les dispositions relatives au futur conseil d'évaluation de l'école pour en faire l'instance produisant la politique d'évaluation de l'éducation nationale. Avec pas moins de quatre entités chargées de cette politique, la fonction d'évaluation paraît dispersée, voire éclatée. Cela contribue à la faiblesse de la diffusion des rapports et des études du ministère et à la faible incidence de cette production, pourtant d'une grande qualité. S'il était adopté, cet amendement permettrait de parachever le renforcement de la fonction d'évaluation prévue par l'article 9. Le conseil d'évaluation de l'école deviendrait ainsi le pilote de la politique d'évaluation du ministère, laquelle serait animée par les services compétents et par ce qui résultera de la fusion des inspections générales.

Je souscris aux modifications adoptées en commission visant à garantir la pleine indépendance du futur conseil d'évaluation de l'école, notamment la capacité des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat à le saisir, dispositions relatives à la composition et aux modalités de nomination de ses membres. Cet amendement vise à apporter des garanties supplémentaires d'indépendance au futur conseil en modifiant sa composition et les modalités de nomination de ses membres, tout en veillant à un équilibre entre autorités de proposition et de nomination des différents collèges, afin que, comme le faisait remarquer la Cour des comptes, le ministère de l'éducation reste totalement responsabilisé sur cet enjeu majeur par son implication au coeur de l'instance. Nous sommes donc à la croisée et des recommandations de la Cour et des débats qui ont eu lieu aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au sein de la commission du Sénat. Je reprends ainsi plusieurs propositions de M. le rapporteur. Tout d'abord, le président de l'instance sera nommé par le Président de la République. En outre, le rôle du Premier ministre, garant du caractère interministériel du conseil d'évaluation de l'école, est renforcé dans la désignation des personnalités qualifiées. Les six personnalités qualifiées seront en effet nommées par le Premier ministre sur désignation de personnalités extérieures au ministère pour la moitié d'entre elles- par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat et par le chancelier de l'Institut de France. Les trois autres personnalités seront proposées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Toujours dans le souci de garantir une plus grande indépendance à l'égard du ministère de l'éducation nationale, il est prévu que l'une des trois personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale soit de nationalité étrangère. Comme proposé par M. le rapporteur, le mandat du président du l'instance et des six personnalités qualifiées sera fixé à six ans. De la sorte, le Parlement sera à l'origine de la désignation de six des douze membres du futur conseil. En effet, outre ses propositions pour deux des six personnalités qualifiées, le nombre de parlementaires n'est pas modifié, le conseil bénéficiant de la présence de deux sénateurs et de deux députés. La pleine association du Parlement aux travaux du conseil sera ainsi garantie. Enfin, comme l'a proposé M. le rapporteur, le nombre de représentants du ministre chargé de l'éducation nationale diminue et est ramené à deux, au lieu de quatre dans le projet initial. Il s'agirait du chef de service de l'Inspection générale-

sur les autres amendements. Cet amendement vise à soumettre la désignation des personnalités qualifiées par les présidents des assemblées à l'avis préalable de la commission permanente compétente de chaque assemblée.

et de la séparation des pouvoirs. Enfin, il ne me paraît pas nécessaire de déterminer avec une telle précision quels seront les représentants du ministre de l'éducation nationale.

d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Nous proposons, par cet amendement, d'ajouter au champ de compétences de l'Opecst une mission qu'il exerce déjà en partie et d'en faire l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques, technologiques et éducatifs.

monsieur le rapporteur,

la pratique ; elle permettrait simplement d'assoir juridiquement des missions qui sont aujourd'hui réalisées par l'Opecst, lequel se verrait ainsi conforté dans son travail d'analyse des politiques générales relatives à la connaissance.

les apprentissages évalués par le personnel éducatif. En 2017, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes rendait publique la première évaluation de la formation initiale et continue des personnels éducatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes, à partir d'une enquête conduite en 2016, soit trois ans après l'adoption de la loi de 2013 et l'inscription de l'égalité entre les filles et les garçons et entre les femmes et les hommes au nombre des valeurs devant être transmises par le service public de l'éducation. Cette évaluation a été particulièrement contrastée. L'offre de formation initiale en matière d'égalité entre les femmes et les hommes est la plupart du temps optionnelle, et peu de modules de formation continue y font référence dans les plans académiques de formation. Il convient donc de réaliser une nouvelle évaluation permettant de mesurer l'effectivité de la formation des élèves à l'égalité entre les filles et les garçons et entre les femmes et les hommes, l'effectivité de la formation initiale des personnels éducatifs à la transmission de ces valeurs aux élèves, quelle que soit la discipline concernée, et l'existence de modules de formation continue

Brulin. Il s'agit de faire en sorte que les enfants instruits à domicile puissent participer aux examens blancs, ce qui leur permettrait de participer aux examens en conditions réelles, et c'est une bonne chose.

reposant sur le libre choix des parents, elle constituerait une contrainte importante et peu prévisible pour les établissements concernés. Avis défavorable sur ces deux amendements. Quel est l'avis

qui feraient le choix de participer aux évaluations organisées à l'échelon national doivent le faire au sein d'un établissement d'enseignement public et que leurs épreuves doivent être corrigées par le personnel enseignant de cet établissement. Il serait dommage que l'article 9 A ait pour effet que, dans certains cas, ces évaluations ne soient pas réalisées et corrigées par les professeurs. Tel n'est pas, en effet, l'esprit de cet article, car, selon les auteurs de l'amendement, la transmission des résultats aux familles leur permettra d'adapter leur projet pédagogique en vue de la maîtrise du socle commun par leur enfant à l'issue de la période d'instruction obligatoire telle que prévue par la loi. Cet amendement a donc pour objet d'instaurer un climat de confiance et de dialogue entre les services de l'éducation nationale et les parents ayant choisi l'instruction à domicile, et de permettre aux élèves instruits à domicile

du Gouvernement ? L'article 9 A du projet de loi, qui est issu d'un amendement parlementaire, confie à l'autorité compétente en matière d'éducation, l'éducation nationale, le soin d'informer les familles des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées à l'échelon national par le ministre de l'éducation nationale. Je ne suis évidemment pas opposé par principe à la présente proposition, mais je pense qu'elle n'a pas sa place dans la loi : il s'agit d'une question d'organisation des services, qui relève donc du pouvoir réglementaire et fera, à ce titre, l'objet de dispositions réglementaires. Cela permettra d'ailleurs d'envisager des dispositifs de mise en oeuvre distincts entre les évaluations en classes de CP et de CE1, d'une part, et les évaluations en classes de sixième et

ne sont pas des composantes universitaires comme les autres ; ce sont avant tout des écoles professionnelles de formation de fonctionnaires de l'État. Il est donc bien normal que l'État employeur indique clairement, y compris dans le choix l'engagement qui est le sien. Nous avions d'ailleurs, dans un rapport dont il faudra peut-être assurer le retirage compte tenu de la fréquence à laquelle nous le citons, bien indiqué qu'il était nécessaire

Cet amendement vise à mieux équilibrer l'année de master 2 : les périodes de stage pratique ne dépasseraient pas un tiers du temps global de formation, selon un rythme plus progressif et donc plus propice

amendement est donc satisfait par l'état actuel du droit. J'en demande le retrait. Concernant l'amendement de M. Ouzoulias, les stages sont un élément essentiel de l'apprentissage du métier d'enseignant.

Faisons confiance aux acteurs de terrain pour établir des maquettes de formation équilibrées au regard des besoins de professionnalisation des futurs enseignants et respectueuses de leur charge de travail globale. Quel est l'avis

futurs enseignants à la prise en charge des élèves en situation de handicap. Cela renvoie à des débats que nous avons eus par ailleurs ; l'objectif est tout à fait louable.

qui est le plus important pour l'amélioration de la qualité du système scolaire, c'est-à-dire la formation des professeurs. J'assume complètement l'idée que cette nomination ne doit pas être laissée au hasard, mais maîtrisée dans le sens de la qualité. d'ores et déjà des directeurs de qualité ; mais cela résulte de processus que je qualifierais d'aléatoires. Au demeurant, les signatures de la ministre de l'enseignement supérieur et du ministre de l'éducation nationale

d'occuper les fonctions de directeur de ces écoles appartient au conseil des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. La disposition visée prévoit une recentralisation de la nomination des directeurs, ce qui ne paraît ni nécessaire ni souhaitable.

cas actuellement, ainsi que la proposition du nom par le conseil d'école, mais dans le cadre du dispositif voulu par le Gouvernement : une audition par un comité des candidats. Nous avons déjà exposé toutes les raisons de notre opposition à une telle réforme : indépendance des instituts du ministère, nécessité de confiance du conseil de l'école dans son directeur ... Je n'insiste donc pas. L'amendement

confrontés à des défis sociaux, comme l'évolution des métiers et des compétences, à des défis stratégiques, notamment celui de la souveraineté numérique appliquée à l'éducation, à des défis démocratiques, en particulier les risques d'aggravation de la manipulation

constate dans tous les secteurs de la société : la formation des formateurs. J'ai d'ailleurs adressé un courrier au Président de la République et au Premier ministre pour que la montée en compétence du numérique de tous nos concitoyens fasse l'objet d'une grande cause nationale. Cet amendement

dans le cadre pédagogique et, plus largement, dans la vie du citoyen, choix des outils. Le deuxième est celui de la connaissance des cultures numériques et des usages : fonctionnement d'internet, connaissance et compréhension des enjeux liés à l'écosystème numérique, notamment le traitement de l'information, la souveraineté des données, l'empreinte numérique, le cyberharcèlement ... Le troisième est celui de l'usage pédagogique de ces outils et ressources numériques : analyse de pratiques pédagogiques innovantes, intégration des technologies numériques dans les enseignements, notamment pour faciliter l'apprentissage et la scolarité des élèves à besoins particuliers. Monsieur le ministre, j'ai bien conscience que

et prévu que, dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées devait tenir compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert. Mais ce simple encouragement n'a pas réellement eu d'effet en pratique. J'avais déposé un amendement visant à inscrire dans la loi la priorité accordée

de l'école de la République, il semble qu'elle n'est pas toujours dispensée dans les écoles. La sensibilisation des futurs professeurs aux enjeux environnementaux permettrait de les inciter à intégrer plus largement les thématiques environnementales dans leurs enseignements. Elle doit également leur permettre de modifier leur propre comportement au quotidien, comportement qui influence celui des élèves. Dans le cadre des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, les futurs professeurs bénéficient déjà de formations de sensibilisation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, de lutte contre les discriminations, de manipulation de l'information, ou encore de scolarisation des élèves en situation de handicap.

Ces deux amendements identiques sont largement complémentaires de l'amendement de M. Maurey que nous avons adopté hier. Il s'agit ici d'inscrire les enjeux liés « au respect et à la protection de l'environnement et à la transition écologique » dans la

langues des outre-mer figurent parmi les soixante-quinze langues régionales ou minoritaires de France. Ces langues, pour la plupart vivantes, restent pour quelques-unes d'entre elles menacées de disparition. Je pense notamment aux langues amérindiennes. Cette vitalité linguistique fait ainsi coexister une pluralité de langues aux côtés du français. Pour cette raison, des approches pédagogiques spécifiques ont été mises en oeuvre, notamment en Guyane avec le déploiement des intervenants en langue maternelle qui effectuent un travail fondamental auprès des enfants allophones. Dans cet esprit, le présent amendement vise à ce que les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation préparent les enseignants aux enjeux du plurilinguisme

un peu plus vagues « d'autres secteurs que l'éducation nationale en qualité d'intervenants extérieurs ». Il serait dommage, par exemple, que l'on ne puisse pas solliciter les personnes du monde associatif.

de contractuels, etc. Concernant les élèves, la continuité pédagogique et la stabilité de leur lieu d'éducation ne sont jamais acquises, alors même qu'un établissement d'éducation prioritaire a pour vocation d'offrir à ses élèves un cadre de nature à pallier les conséquences des inégalités socio-économiques par « un renforcement de l'action pédagogique et éducative ».

La corrélation entre l'expérience et le turnover des enseignants nous semble révélatrice : il s'agit bien évidemment non pas d'insinuer que les enseignants ne sont pas assez compétents, mais bien

car, au bout du compte, un professeur est seul face à ses élèves la majorité du temps. Il faut qu'il y soit préparé. Si être professeur, c'est exercer le plus beau métier du monde, c'est aussi exercer un métier prenant

monde. Quel est l'avis de la commission ?

initiale continuée, s'inscrivant dans la durée. On ne peut pas tout apprendre dans les Espé avant la titularisation. Prenons d'ailleurs garde à ne pas trop charger la barque de cette formation initiale, sous peine d'éparpillement et de dispersion.

discussions qui ont lieu avec les organisations syndicales et l'ensemble des partenaires, puisque le référentiel de formation va prévoir que 10 % du temps sera consacré aux spécificités du territoire. Cet

Toutefois, en respectant les contraintes de l'article 40 de la Constitution que je n'ignore pas, je ne pouvais pas aborder autrement que par ce biais la question de la visite médicale des personnels enseignants, qui me paraît au demeurant extrêmement problématique, ce qui justifie à mes yeux une expertise sur sa généralisation. En pratique, les professeurs des écoles ne voient le médecin du travail qu'une fois au cours de leur vie professionnelle, au moment de leur titularisation, alors qu'une visite régulière serait requise, car ils sont en contact permanent avec les enfants. La visite médicale permet de s'assurer du maintien de l'aptitude de l'intéressé au poste de travail qu'il occupe et de dépister les maladies dont il pourrait être atteint. Il me paraît donc justifié de rétablir l'article 13 demandant un rapport sur la faisabilité de la généralisation de la visite médicale pour les personnels enseignants tout au long de leur carrière, à moins que M. le ministre ne soit porteur du message auprès de Mme Buzyn,

collègue. Tous les agents de la fonction publique d'État devraient en principe bénéficier d'un examen médical d'aptitude lors de leur prise de poste, puis en cours de carrière à l'occasion de chaque changement. En outre, ils sont tenus de se soumettre à un examen médical par le médecin de prévention tous les cinq ans. Les obligations en matière de médecine de prévention existent donc et s'appliquent au ministère de l'éducation nationale.

découvrir et apprendre progressivement et sans pression ce métier le cumul d'une rémunération et d'une bourse d'études. Par ce biais, l'objectif est, d'une part, de renforcer l'attractivité du métier d'enseignant à travers une accession plus aisée des jeunes issus des classes populaires à une carrière de professeur et, d'autre part, de permettre aux enseignants en devenir d'acquérir des compétences pédagogiques pratiques. Néanmoins, vous le comprendrez aisément, monsieur le ministre, plusieurs collègues et moi-même avons un certain nombre de questions sur ce nouveau mode de recrutement. Ainsi, les assistants d'éducation se verraient octroyer un salaire compris entre 893 et 980 euros par mois dès leur deuxième année de licence, à condition de préparer les concours de professeur des écoles, de collège ou de lycée. Mais est-ce un salaire brut

pouvez-vous certifier, devant la Haute Assemblée, que ce mode de prérecrutement n'a pas vocation, à court, à moyen ou à long terme, à pallier, à coût réduit, les difficultés de recrutement et de remplacement des enseignants, ce qui risquerait d'accélérer la dévalorisation des vocations éducatives ? L'amendement

Le dispositif, s'il était bien encadré, permettrait aux jeunes de se préparer au métier d'enseignant et, éventuellement, être source d'attractivité pour la carrière. Mais il faut être très prudent : comme on l'a dit, se retrouver tout seul face à une classe est très dur

dans un nécessaire parcours de préprofessionnalisation dès leur deuxième année de licence. C'est pourquoi la commission ne souhaite pas la suppression de cet article.

Nous savons que ces IPES avaient mille vertus pour le système scolaire, d'abord, d'un point de vue social, pour les personnes concernées, mais aussi pour le système lui-même, puisqu'ils contribuaient à encourager les vocations,

légèrement supérieure à 700 euros nets, monsieur le sénateur, cumulable avec une bourse, ce qui pour certains étudiants pourrait représenter entre 900 et 1 000 euros au total. Je vous le dis très franchement : si j'étais un étudiant

de grandes vertus sociales : d'abord, elle vise l'élargissement sociologique du vivier de nos futurs professeurs, alors que nous savons tous que la mastérisation a eu

nous considérons que, du point de vue des assistants d'éducation, notamment lorsqu'ils seront en M1, les missions d'enseignement, sous la responsabilité de leur tuteur, peuvent être intéressantes en termes de préprofessionnalisation préprofessionnalisation et de validation de leur projet professionnel. Il serait dommage de les priver d'une telle expérience. L'amendement n° 438 rectifié vise un référentiel des missions des assistants d'éducation. Je

des futurs enseignants, qui auront choisi de passer par la préprofessionnalisation. En effet, afin d'améliorer l'insertion des élèves en situation de handicap au coeur des classes traditionnelles, il pourrait être précieux de permettre aux futurs enseignants de mieux appréhender et comprendre les difficultés spécifiques de ces enfants. Aussi pourrait-il être pertinent et formateur d'inclure dans le cursus des futurs professeurs, notamment des assistants d'éducation concernés par la préprofessionnalisation, une période consacrée exclusivement à l'accompagnement d'élèves handicapés. l'apprenti enseignant effectuerait alors la même mission que les AESH, afin de bien intégrer les attentes et besoins de l'élève sous sa responsabilité. L'expérience ainsi acquise serait évidemment utile aux futurs maîtres lorsqu'ils devront gérer des effectifs comprenant

Certes, votre amendement part d'une très bonne intention : former les futurs enseignants aux difficultés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Je pense quand même que, au cours des périodes d'observation en classe, les assistants d'éducation auront l'occasion de croiser des AESH, de prendre connaissance de la réalité de leur métier, et de partager avec eux.

Laborde. À l'occasion d'une question orale au Sénat, le 12 février dernier, mon collègue Jean-Yves Roux vous avez alerté, monsieur le ministre, sur les difficultés des collèges et lycées ruraux, qui peinent à recruter des assistants d'éducation. 7,3 % des jeunes ruraux possèdent un diplôme universitaire de deuxième ou troisième cycle universitaire, contre 15,4 % des jeunes des aires urbaines. les assistants d'éducation sont traditionnellement recrutés parmi les étudiants boursiers. Or les jeunes gens ou jeunes filles susceptibles d'être intéressés par ces métiers étudient trop loin des établissements recrutant en milieu rural. Leur temps de déplacement et leur facture d'essence, assortis de salaires faibles et d'un temps de travail décousu, constituent des freins importants. Nous insistons donc sur la nécessité d'introduire de la souplesse pour recruter ces assistants d'éducation, jeunes ou moins jeunes. Par ailleurs, monsieur le ministre, en réponse à cette question orale, vous aviez envisagé une réforme plus globale du recrutement des AESH et assistants d'éducation dans ces secteurs, afin de compléter les salaires, d'assurer un véritable statut d'accompagnement scolaire, pour augmenter le niveau de formation et de compétences et limiter les déplacements. Le projet de loi prévoit de recruter, parmi les assistants d'éducation, des jeunes qui poursuivent un cursus menant à un métier d'enseignant.

de ces assistants candidats vers les zones sous-dotées, en ouvrant la possibilité d'indemnisations renforcées. Quel

Mme la présidente de la commission.

Madame Cartron,

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est ouvert.

en matière de réussite scolaire et éducative. » Si des efforts ont été consentis, à raison, pour renforcer l'école dans certains quartiers, les écoles rurales rencontrent aussi des difficultés qui ne doivent pas être minimisées, notamment en matière de recrutement des professeurs. Afin de répondre aux défis de l'affectation des enseignants dans les territoires les plus difficiles, ruraux comme urbains, en zone REP, la commission a introduit l'affectation sur contrat de mission, par lequel l'affectation de l'enseignant procède d'un engagement conclu avec le recteur, pour une durée déterminée et pouvant s'accompagner de conditions particulières. Ce contrat est un moyen incitatif de lutter contre la désertification scolaire dans les zones dites difficiles. En vue de garantir une meilleure efficacité de ce dispositif, il est nécessaire de préciser, avant de s'en remettre aux modalités fixées par décret, que ces contrats de mission bénéficieront prioritairement aux zones d'éducation prioritaire- REP et REP+ -et aux écoles situées en zones hyper-rurales, où la désertification scolaire est une réalité. est le sens de cet amendement de précision. Max Brisson et Françoise Laborde avaient, dans le cadre de leur rapport, suggéré de permettre aux recteurs de compenser, par des primes modulées, les différences d'attractivité entre les postes, non seulement en REP et REP+,

a été créé par le décret du 1 février 2017. La mission de ces psychologues dépasse largement le cadre du dépistage et porte sur le rapport à la réussite scolaire de tous les enfants et adolescents, le suivi individualisé et l'accompagnement à l'élaboration de leur projet d'avenir en lien avec les parents. L'ancrage psychopédagogique des psychologues de l'éducation nationale est donc une caractéristique de la fonction, depuis sa création. Les textes réglementaires relatifs au nouveau statut donnent de nombreux exemples de cette complémentarité à rechercher avec les équipes pédagogiques et les familles. Ces professionnels

Monsieur le rapporteur,

Je l'ai dit à M. le rapporteur en commission : je n'arrive toujours pas à voir le lien entre cette disposition et le présent texte sur l'école. J'ai bien l'impression qu'il s'agit là d'un cavalier législatif.

de recherche. Le texte qu'elle présentera prochainement devant le Parlement serait un meilleur véhicule législatif pour cette disposition.

Sur le fond, cet article prévoit que l'examen des conditions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs relève du conseil académique siégeant en formation restreinte aux seuls représentants élus de ces derniers, des chercheurs des chercheurs et des personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui-ci. Le nouveau dispositif ouvre la possibilité que les statuts d'un établissement dérogent à cette règle et au président ou au directeur de ce conseil de présider ce dernier. Dans la pratique, de nombreux conseils académiques, même lorsqu'ils siègent en formation restreinte, sont d'ores et déjà présidés par le président ou le directeur de l'université. Il ne semble pas utile d'inscrire dans la loi une disposition qui, par nature, marque un recul pour l'indépendance des enseignants-chercheurs.

présenter l'amendement n° 78 rectifié . Le but visé à travers cet amendement est de rester dans le cadre juridique tel qu'il est défini depuis 2015. Il convient de souligner que celui-ci résulte d'un dialogue social auquel les infirmiers scolaires restent attachés. Il s'agit donc d'une demande formulée par de nombreux professionnels, qui ne souhaitent pas revenir en arrière. Tout d'abord, il est nécessaire de préciser que le droit actuel définit le champ de la promotion de la santé à l'école selon sept axes environnement scolaire, programme d'éducation à la santé, participation à la politique sanitaire nationale, coordination avec la PMI, réalisation d'examens de santé et détection précoce des troubles pouvant entraver la scolarité, accueil et suivi individuel des élèves, veille épidémiologique. En outre, le présent article prévoit que la santé à l'école sera gérée en « équipes pluriprofessionnelles ». Or il est important de souligner que cette rédaction revient à passer d'une démarche globale holistique, telle que définie par la loi d'orientation et de programmation pour

L'article 16 pouvait paraître bien anodin : il prévoit que les médecins, les infirmiers et les assistants sociaux de l'éducation nationale travaillent en équipes pluriprofessionnelles. Mais il a suscité un très grand émoi, les infirmiers notamment y voyant la remise en cause du cadre de travail établi en 2015. J'ai rencontré l'ensemble des syndicats des personnels concernés et je dois avouer que je n'ai

Les médecins scolaires, comme tous les médecins inscrits à l'ordre des médecins, ont un droit de prescription qui fait intégralement partie de leurs missions. L'article 16 ne vise qu'à en sécuriser le principe. Demande de retrait ou avis défavorable.

Le premier alinéa tend ainsi à rendre effectif le remboursement des prescriptions des actes diagnostiques et préventifs des médecins de l'éducation nationale, particulièrement ceux qui sont en lien avec la scolarité de l'enfant. Cette disposition permettra de faciliter l'accès aux soins, de réduire les inégalités territoriales et de renforcer la prévention. Ce dispositif s'avère être également source d'économies en ce qu'il évite les consultations uniquement justifiées par le besoin de prescription. Les actes concernés seront des actes ou des produits préventifs, tels qu'un bilan orthophonique ou orthoptique, un vaccin, une contraception. Un décret en précisera la liste. Plusieurs rapports sur la médecine scolaire ont préconisé cette mesure, qui est également inscrite au plan national de santé publique 2019 dans le cadre de la stratégie nationale de santé 2018-2022. vise également à apporter des précisions et des améliorations rédactionnelles. Par exemple, la formulation « ces actes et produits sont remboursés par les caisses d'assurance maladie dans les conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale » est préférable à la précédente rédaction, plus ambiguë, qui pouvait laisser entendre que des actes ou produits non remboursés

la santé publique. Le second alinéa de l'amendement a pour objet de sécuriser juridiquement l'administration aux élèves ou aux étudiants, par les infirmiers de l'éducation nationale, de médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire, dont la liste sera fixée par décret. Pratiquée sauf indication contraire d'un médecin ou des responsables légaux de l'enfant, l'administration ainsi encadrée de certains médicaments permet un retour rapide en classe ou permet de soulager l'élève dans l'attente d'une prise en charge adaptée. De plus, cette administration par un professionnel de santé permet de limiter les risques d'automédication des élèves. Enfin, cet alinéa sécurise juridiquement l'administration par les infirmiers de l'éducation nationale de médicaments soumis à prescription médicale obligatoire dans le cadre des protocoles, en particulier le protocole national de soins et d'urgence élaboré par le ministère de l'éducation nationale avec le ministère chargé de la santé. sécuriser utilement ces activités importantes au quotidien pour la santé et la scolarité des élèves, dans le respect du droit de s'y opposer que détiennent évidemment les responsables légaux de l'enfant. C'est donc un amendement pragmatique.

Après confirmation de M. le rapporteur, je retirerai l'amendement

tout au moins. Cela devrait permettre de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Il s'agit également d'une mesure d'économie à l'échelle familiale, mais aussi nationale. Néanmoins, quitte à offrir cette possibilité aux médecins scolaires, il me semble que nous aurions dû en faire autant pour les infirmiers et infirmières scolaires. Pourquoi ? Je rappelle que les infirmiers et infirmières de l'éducation nationale sont les conseillers en santé des équipes éducatives et pédagogiques, des chefs d'établissement, des directeurs d'école, des inspecteurs d'académie-directeurs Dans leur cadre spécifique d'exercice, les infirmiers et infirmières de l'éducation nationale ont également recours à des dispositifs et réalisent aussi des actes visant la prévention, la détection des la détection des troubles de la santé, l'amélioration de l'accès à la contraception et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles. Ils rencontrent dès lors quotidiennement les mêmes difficultés que les médecins scolaires, notamment avec les caisses d'assurance maladie. C'est pourquoi il me semble qu'aurait dû être organisée en amont une rencontre entre le ministère, les médecins scolaires et les infirmiers et infirmières scolaires, afin d'aboutir à un consensus sur le sujet. N'oublions pas que ces derniers sont très souvent le professionnel de santé

est à M. le ministre. Cet amendement vise à remplacer l'habilitation- supprimée par la commission -du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer la gouvernance des services déconcentrés des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse, et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

tenant compte des spécificités des territoires qu'il administre. C'est là une étape importante qui doit nous permettre de mettre en place cette organisation territoriale dont j'ai déjà eu l'occasion de parler lors de précédents débats précédents débats et de tirer les conséquences de la réforme régionale en vue d'une meilleure adéquation entre l'organisation du système éducatif et les régions-

que cette structure ne fonctionne pas très bien, alors qu'elle pourrait rendre de très grands services, notamment dans le cadre de la relation indispensable entre les services départementaux de l'éducation nationale et les élus, les administrés

pour la gouvernance de notre école. Avis défavorable.

d'enseignement. En effet, il est essentiel de garder le cadre d'un établissement dont le conseil décisionnaire est présidé par un membre présent tous les jours dans les lieux, et donc plus proche de la réalité du terrain qu'une

que cette règle qui fonctionne bien dans les lycées professionnels ne peut pas être appliquée sans négociation non seulement avec les personnels de direction, mais aussi avec les enseignants et les parents d'élèves, qui font partie intégrante des conseils d'administration. La parole

qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs

Le scrutin est ouvert.

assurée par les établissements publics locaux d'enseignement, ou EPLE. Actuellement, plusieurs EPLE peuvent passer une convention entre eux pour mutualiser la paie des agents qu'ils recrutent- assistants d'éducation, AESH, contrats aidés, etc. Toutefois, le périmètre de ces mutualisations résulte d'accords entre EPLE et certaines rémunérations ne sont pas intégrées au dispositif de mutualisation mis en place, notamment les paies ponctuelles, les rémunérations des personnes qui participent aux classes de découverte, les vacations diverses, etc. Or l'arrivée de la déclaration sociale nominative, la DSN, dans la fonction publique va nécessiter que tous les agents rémunérés soient déclarés tous les mois. Pour faciliter le travail des gestionnaires des établissements, le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse est en train de développer un logiciel de paie pour les EPLE, qui s'appelle OPER@. Il facilitera les démarches de mutualisation de la paie entre les EPLE. Pour mener à bien ces évolutions, il est nécessaire que toutes les paies effectuées par les EPLE soient recensées et fiabilisées dans un cadre automatisé. Cet amendement a donc pour objet de confier à l'État l'organisation de la mutualisation de la paie des EPLE, afin que les périmètres de mutualisation soient homogènes et couvrent l'intégralité des rémunérations versées par les EPLE.

L'article L. 131-13 issu de la loi Égalité et citoyenneté a instauré un droit d'accès à la restauration scolaire pour tous les enfants scolarisés. Cet amendement permet de concilier ce droit d'accès avec les capacités réelles des communes. Avis favorable. Quel est ? Je comprends l'inspiration des auteurs de cet amendement. Néanmoins, nous menons une politique volontariste pour la cantine, vous le savez, notamment avec les différentes opérations

qu'elles sont réalisables en pratique. Je pense que nous n'enverrions pas un bon signal en revenant en arrière par rapport à ce que la loi a établi. Je m'en remets

dans une ville comme Saint-Laurent-du-Maroni pour répondre à la pression démographique. Face à cette situation, notre commission a adopté une expérimentation permettant de déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction et de commande publique. publique. Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine les règles qui peuvent faire l'objet de cette expérimentation. Or, le droit de la commande publique relevant du domaine de la loi, seule une disposition législative peut permettre des dérogations. Ainsi, le seul renvoi à un décret serait considéré comme une incompétence négative du législateur. À cet égard, le Conseil constitutionnel censure les dispositions législatives reportant sur l'autorité administrative le soin de fixer des règles dont la détermination relève du domaine de la loi. C'est pourquoi le présent amendement récrit l'article de manière à préciser que les dispositions relatives à la procédure de conception-réalisation peuvent faire l'objet de dérogations. Si, en principe, le recours à cette procédure n'est possible, pour les acheteurs, que dans des hypothèses limitativement énumérées, le législateur a déjà autorisé un libre recours à ces marchés. C'est le cas de l'article 69 de la loi ÉLAN qui autorise, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2022, les CROUS à recourir librement aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements. Autoriser, en Guyane et à Mayotte, un libre recours aux marchés publics de conception-réalisation pour la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles d'enseignement public, répond à une demande forte des élus. Cela permettra d'accélérer le processus de passation des marchés, la réalisation des travaux et, à terme, de scolariser de nombreux enfants. L'enjeu est important pour ces territoires. Quel est l'avis de la commission ? Les auteurs de cet amendement proposent une nouvelle rédaction de l'article 21 adopté par la commission pour la Guyane et Mayotte. Avis favorable. monsieur le ministre,

dans certaines collectivités d'outre-mer. Cependant, si cette procédure se justifie pleinement pour certaines dispositions, il en est d'autres pour lesquelles il est regrettable de perdre de longs mois pour les rendre applicables. Il est donc proposé que certains articles du présent texte soient rendus directement applicables à Wallis-et-Futuna sans attendre la ratification d'une ordonnance.

Si la présente loi ne prévoit pas expressément l'application de certaines de ses dispositions dans les îles Wallis et Futuna, c'est parce que nous avons fait le choix de procéder par voie d'ordonnance à l'actualisation des dispositions de nature législative du code de l'éducation relatives à l'outre-mer-

procéder par ordonnance afin de conduire ce travail avec rigueur et méthode et d'éviter toute erreur. Il ne me paraît donc pas approprié de procéder à une extension partielle d'une partie du projet de loi à une seule des collectivités d'outre-mer- c'est d'ailleurs ce que

Nos élèves sont pénalisés par l'enclavement de notre territoire, avec tout ce que cela implique. Beaucoup d'entre eux se retrouvent, sinon en situation d'échec scolaire, du moins en très grande difficulté. Des ordonnances vont être prises : il faut qu'elles le soient rapidement et en concertation avec les élus et les services du territoire, qui connaissent bien la situation. L'amendement

monsieur le ministre, mes chers collègues, hier, j'ai évoqué la situation matérielle catastrophique que nous subissons, notamment en raison de dégradations du bâti. J'ai accepté à contrecoeur de retirer mon amendement, mais je voudrais revenir sur le problème. Qu'un plafond se soit effondré du fait de malfaçons, de dégradations, c'est un désastre. Imaginez s'il y avait eu des victimes pendant un cours ... À vouloir faire des économies, nous mettons en danger la vie des élèves et des enseignants. Je rappelle de nouveau que les dépenses liées à l'enseignement seront à Wallis-et-Futuna intégralement à la charge de l'État. Il y a donc urgence ! Des ordonnances, c'est bien, mais c'est long. Il faut réfléchir et agir vite. Une réflexion doit être menée sur la prise en charge des dépenses qui, actuellement, ont été confiées au ministère des outre-mer. Peut-être faut-il revenir à une gestion directe par vos services, monsieur le ministre ? Autre point : l'enseignement primaire est confié par délégation à la mission catholique. À la suite d'une rencontre du président de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna avec votre directeur de cabinet, il a été convenu de consolider juridiquement l'assise de la convention de concession de l'enseignement primaire. Je souhaiterais savoir où nous en sommes et si les ordonnances prévues par l'habilitation résultant de cet article régleront ce point. Je suis saisi

législative, ainsi qu'à l'évolution du statut de Mayotte ; extension de l'application de certaines dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et Wallis-et-Futuna. Le Parlement ne peut pas signer un chèque en blanc au Gouvernement pour lui permettre, sans aucune indication, d'étendre de nombreuses dispositions du code de l'éducation à de très nombreux territoires d'outre-mer. Les élus concernés souhaitent pouvoir débattre de ces extensions.

Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Par souci de clarté et de lisibilité de la norme, l'ordonnance que le Gouvernement est autorisé à prendre pour l'actualisation des dispositions législatives du code de l'éducation relatives aux collectivités d'outre-mer répartira dans des divisions nouvelles les articles relevant respectivement de la compétence de l'État, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française et il en résultera une nouvelle numérotation des articles concernés. La nouvelle répartition des articles permettra d'identifier plus aisément les compétences respectives de l'État, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française en matière d'éducation. Cet amendement est donc purement formel et rédactionnel.

Cet amendement tend à supprimer l'article 23 introduit par la commission, sur l'initiative de notre collègue Laurent Lafon, pour autoriser les établissements privés à dispenser des formations en alternance. La loi Pénicaud avait autorisé les établissements publics d'enseignement à dispenser des formations en alternance.

Mme Samia Ghali. Cet amendement vise à fixer, par décret en Conseil d'État, le taux d'encadrement minimal pour l'accueil des élèves pendant les temps de pause. Ce décret respectera les normes Afnor : un pour trente enfants en élémentaire. Ce décret a pour but de faire respecter par les écoles sous contrat éducatif local avec l'État un taux d'encadrement permettant d'assurer la sécurité des élèves, ainsi que des conditions de travail décentes pour les encadrants.

régulièrement avec le recteur de Marseille, qui lui-même parle évidemment avec les collectivités locales, et notamment la municipalité. Nous avons sans doute à progresser sur certains cas,

Je ne ferai pas de commentaire sur le fond. Cet amendement vise à rétablir l'article 24 qui prévoyait un rapport sur l'état du bâti des écoles marseillaises et que la commission avait supprimé. Je propose à nos collègues

Le scrutin est ouvert.

liés à l'exposition des enfants et de la communauté éducative à l'amiante et aux polluants de l'air intérieur, notamment le formaldéhyde, présent dans les établissements scolaires.

Il est donc déraisonnable de prévoir l'applicabilité de la majeure partie de ce texte dès la rentrée de septembre 2019 : par pragmatisme, nous demandons son report à la rentrée de

à nos côtés pendant ces jours denses, mais passionnants.

nous avons, nous aussi, nos divergences et nos convergences. Parfois, les divergences s'estompent, mais il est rare que les convergences disparaissent. Je suis très heureux de tous les progrès que nous avons faits au cours de ce processus